par les articles 30, 35 et 39-1 du code de procédure pénale. Surtout, il ne paraît pas justifié de prévoir que ces rapports devront être adressés par les procureurs au Parlement. Cela serait inutile, puisque ces rapports sont déjà rendus publics, mais cela me semble en outre poser un problème constitutionnel au regard de la séparation des pouvoirs. C'est en effet au Gouvernement, et, en l'espèce, au ministre de la justice, garde des sceaux, de rendre compte devant le Parlement de sa politique pénale, et non pas aux différentes autorités judiciaires. Au reste, l'article 39-1 du code précité prévoit que chaque procureur de la République adresse au procureur général un rapport de politique pénale ; l'article 35 prévoit que le procureur général adresse une synthèse de ces rapports au garde des sceaux ; l'article 30 prévoit que le garde des sceaux, au vu de ces rapports, élabore un rapport annuel sur l'application de la politique pénale sur l'ensemble du territoire de la République. En outre, l'article 30 précise que ce rapport annuel est transmis au Parlement et qu'il peut donner lieu à un débat devant l'Assemblée nationale et devant

Monsieur Bigot, il appartient au garde des sceaux de faire la synthèse de ces rapports locaux et de vous la présenter. C'est le rôle du garde des sceaux, et c'est ce que je ferai

téléphone sans contact, qui est aujourd'hui un succès national. Or ce dispositif s'est développé à partir d'échanges avec le procureur de la République de Strasbourg au sein du conseil intercommunal de prévention de la délinquance, lorsque j'étais président de la communauté urbaine. Le procureur demandait

Ils se retrouvent pour commettre leurs méfaits dans nos métropoles ou dans notre environnement, puis ils se retrouvent dans les maisons d'arrêt du secteur. Nous avons donc besoin de travailler ensemble. Les magistrats n'y sont pas toujours prêts, et je pense qu'il faut les y forcer un peu. Tel est le sens de cet amendement ; si ce rapport existe

Le suivi socio-judiciaire a été institué par la loi du 17 juin 1998, présentée par Élisabeth Guigou, relative à la répression des infractions sexuelles. à l'origine pour les seules infractions sexuelles ou pour les infractions mettant en évidence la perversion de leur auteur, y compris le meurtre avec viol, torture ou acte de barbarie, le suivi socio-judiciaire a été étendu en décembre 2005 à tous les meurtres, aux enlèvements et aux incendies volontaires.

qui ont pu être commises dans des circonstances faisant apparaître chez leur auteur des troubles du comportement, principalement de nature sexuelle, susceptibles de faire l'objet d'un traitement médical, alors même que la dimension sexuelle de ce comportement n'apparaît pas dans la qualification juridique C'est pour la même raison que, en 2007, le suivi socio-judiciaire a été étendu aux violences au sein du couple ou commises par un ascendant sur mineur.

qu'aucune des contributions produites ni aucune des personnes auditionnées n'a évoqué l'extension de la peine de suivi socio-judiciaire ». Une telle généralisation aboutirait d'ailleurs à une aggravation sans doute disproportionnée de la répression, puisque le suivi socio-judiciaire s'ajoute à la peine privative de liberté prononcée. cette extension me semble inutile pour empêcher les sorties sèches. Celles-ci peuvent déjà être évitées dans la majorité des cas grâce aux aménagements de peine, aux libérations conditionnelles et suivi post-peine et, dans les cas les plus graves, à la surveillance judiciaire ou à la surveillance de sûreté. L'amélioration de la libération sous contrainte, telle qu'elle est proposée par le Gouvernement, qui facilitera les aménagements en fin de peine, est également de nature à éviter les sorties sèches. Pour toutes ces raisons, je vous demande de supprimer l'article 45 , tel qu'il a été élaboré par la commission.

contre ces sorties en multipliant les aménagements automatiques de peine. Elle préfère au contraire accompagner la peine d'emprisonnement soit d'une peine de probation soit d'une peine complémentaire du suivi socio-judiciaire. Il s'agit certes d'une aggravation de la répression, nous en sommes d'accord, mais qui est totalement assumée et qui permettra d'assurer un réel contrôle

de dire que la proposition de Mme la garde des sceaux est plus exacte, parce que la libération sous contrainte permet à l'administration pénitentiaire de

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec celui qui tendait à élargir le périmètre possible d'un PSE mobile. Il vise à réduire les seuils prévus aux articles 131-36-10 et 131-36-12-1 du code pénal dans le cadre du suivi socio-judiciaire. L'article 731-1 du code de procédure pénale dispose que la personne condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une libération conditionnelle. Il convient d'abaisser ce seuil à cinq ans.

transformant le sursis avec mise à l'épreuve, ou SME, en sursis probatoire pouvant comporter, si la personnalité du condamné le justifie, un suivi individualisé, renforcé, pluridisciplinaire et évolutif fondé sur des évaluations régulières du condamné. Sur le fond, messieurs les rapporteurs, monsieur le président, je crois que nous partageons le même objectif : nous souhaitons disposer d'une mesure efficace qui permette de développer la probation,

pénale, intellectuellement très intéressante en ce qu'elle instituait une peine autonome de probation, n'a été que très peu

la durée de l'emprisonnement encouru par le condamné qui ne respecterait pas ses obligations. Finalement, cette peine de probation que vous prétendez autonome est forcément référencée à l'emprisonnement, puisque la personne qui ne qui ne satisferait pas aux obligations qui y sont liées retournera en prison. Il n'est donc pas intellectuellement correct de dire que la peine de probation est déconnectée de l'emprisonnement. Elle ne l'est pas moins qu'une peine d'emprisonnement

que certains condamnés fassent l'objet d'une mesure de probation renforcée, individualisée et évolutive. Il me semble toutefois que le texte issu des travaux de votre commission est plus complexe, moins lisible et moins efficace que celui que je soutiens. que celui que je soutiens. Prenons l'exemple d'une personne condamnée en récidive pour des faits de violences au sein d'un couple. Avec le sursis probatoire, le tribunal peut prononcer une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans assortis d'un sursis probatoire renforcé. La personne effectue donc une peine de deux ans d'emprisonnement et, à sa libération, fait l'objet

Pour toutes ces raisons, et puisque nous visons le même but, je vous propose d'adopter l'amendement présenté par le Gouvernement et, bien sûr, de poursuivre le travail d'amélioration du texte au cours de la navette.

Par coordination avec l'amendement que nous avons défendu à ce dernier article, cet amendement vise à incorporer, dans le code de procédure pénale, le régime de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique. Dans la lignée de nos précédentes interventions, nous défendons le principe de l'autonomisation de cette peine, dont l'application favorisera les possibilités de réinsertion, tendra à endiguer le phénomène endémique de la surpopulation carcérale, luttera contre les cas de récidive et diminuera l'incidence budgétaire de notre politique pénale.

le soin d'apprécier si une libération conditionnelle est, ou non, possible, sans nécessairement rigidifier la loi de façon excessive.

de vote. Le groupe socialiste suivra la position du Gouvernement et s'opposera à cet amendement. Il faut bien comprendre que la façon dont se déroule une peine est souvent fonction de la possibilité ou non de bénéficier de mesures d'accompagnement ou de libération. Renoncer à ce

le principe selon lequel la libération sous contrainte doit être ordonnée lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir- sauf bien sûr si cela se révèle impossible au regard des exigences de l'article 707 du code de procédure pénale, qui fixe les objectifs de l'exécution des peines, notamment la nécessité de prévenir la récidive. Cette inversion du principe qui fait de la libération sous contrainte la règle, et de son refus, l'exception, vise selon moi un double objectif

de la peine l'examen automatique de la situation des personnes condamnées exécutant une peine inférieure ou égale à cinq ans dans le cadre du dispositif dit « de la libération sous contrainte », aujourd'hui prévu aux deux tiers de la peine. Ce dispositif rogne en effet Ce dispositif rogne en effet de façon trop importante le quantum de peines déjà presque amputées de moitié par le jeu des crédits de réduction supplémentaires, et parfois même exceptionnels, de peine. Décaler au dernier quart

Les auteurs de cet amendement souhaitent introduire un critère de risque de trouble à l'ordre public pouvant fonder le rejet d'une demande d'aménagement, dans une logique plus aboutie d'individualisation des peines.

qui prévoyait que les derniers mois des peines de moins de cinq ans s'exécuteraient sous forme de surveillance électronique, sauf impossibilité, refus du condamné ou risque de récidive. Son caractère en principe automatique, sans décision du JAP, le juge de l'application des peines,

une libération avec surveillance électronique. Il me semble donc que le rétablissement de la SEFIP ancien modèle ne présente guère d'intérêt pratique pour prévenir les sorties sèches. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable

Mme Pascale Gruny. Cet amendement a pour objet qu'aucune libération conditionnelle ne puisse être étudiée avant que le condamné ait effectué au moins les deux tiers de sa peine.

de famille. Il me semble que repousser aux deux tiers de la peine la possibilité de libération d'un détenu qui présente un ou plusieurs de ces différents critères serait contraire à l'objectif de lutte contre la récidive. Le Gouvernement

Les méthodes de déradicalisation mises en place peinent encore à obtenir des résultats satisfaisants. Les détenus condamnés pour des faits de terrorisme présentent pour un certain nombre d'entre eux des risques importants de récidive. Dans de telles situations, la peine de prison trouve son utilité essentiellement dans son rôle de neutralisation. Ainsi un régime spécial d'exécution des peines doit-il être réservé à ce type de détenus, particulièrement dangereux, à l'image de ce qui peut exister en Italie,

Monsieur le rapporteur,

Monsieur le rapporteur,

simplifie et uniformise le traitement des requêtes post-sentencielles. Il prévoit notamment que les décisions de confusion de peines pourront être prises à juge unique, par la modification du dernier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale. Certes, une décision de renvoi vers la formation collégiale est toujours possible, en première instance comme en appel, mais elle risque d'être peu utilisée.

Par cet amendement, il s'agit de rétablir la possibilité pour la commission de l'application des peines de délibérer par voie dématérialisée. telle mesure répond à des observations formulées par les praticiens du terrain. Je le rappelle, la commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines. Elle comprend le procureur, le chef d'établissement pénitentiaire, des membres du personnel de surveillance et des personnels d'insertion et de probation. Sur certains points, il est parfois plus aisé de délibérer par voie dématérialisée. Bien évidemment, cela ne pourra être possible que pour donner des avis qui ne nécessitent pas la réunion physique de l'ensemble des membres de la commission. Si une telle réunion est justifiée, elle se tiendra, la loi ne prévoyant qu'une simple faculté. Selon moi, on ne peut pas refuser de façon systématique les simplifications permises par la dématérialisation.

un amendement visant à supprimer la possibilité prévue par le projet de loi de dématérialiser les échanges lors des commissions de l'application des peines. Ces commissions sont aujourd'hui des instances donnant lieu à des débats parfois intenses entre la direction de l'établissement pénitentiaire, le procureur de la République, le juge de l'application des peines et le service d'insertion et de probation. Nous pensons que la réunion physique de ces personnes est utile. La dématérialisation pose tout de même problème, dans la mesure où il s'agit de prendre des mesures extrêmement importantes concernant les détenus.

garde des sceaux. Cet amendement vise à rétablir les dispositions permettant au chef d'établissement pénitentiaire d'accorder des permissions de sortir lorsqu'une première permission de sortir a été accordée par le juge de l'application des peines, peines, sauf si ce magistrat s'y oppose. Le texte, qui est équilibré, simplifie vraiment la mise en oeuvre des permissions de sortir, tout en permettant au juge de conserver, s'il le souhaite, ses prérogatives en cette matière.

d'une agence nationale de l'exécution des peines, destinée à centraliser les demandes d'exécution des peines présentant une dimension internationale. Cette dernière serait censée constituer un point de contact unique pour les questions complexes d'exécution des peines. Selon moi, la nécessité d'une telle entité n'est pas démontrée. En effet, aucun élément statistique ne précise quel serait le nombre de ces dossiers complexes. De plus, les missions qui seraient confiées à cette agence sont aujourd'hui déjà exercées par les services de mon ministère. Ces derniers assurent effet un soutien opérationnel en matière d'entraide pénale internationale, dans le cadre d'une permanence quotidienne. Ils répondent aux demandes d'analyses juridiques formées par les juridictions pour des situations individuelles anonymisées.

pour simplifier la procédure de reconnaissance des peines privatives de liberté au sein de l'Union européenne. Ajouter un nouvel acteur par le biais de cette agence ne ferait que complexifier les référents et nuirait en réalité à la bonne exécution des décisions, notamment en matière de confiscation,

Nous avons, dans le cadre de la préparation de ce texte, rencontré magistrats, juges du siège, procureurs de la République et juges de l'application des peines. Leurs propos ont régulièrement fait état à la fois de la complexité de notre système et,

vous venez de nous expliquer que votre ministère fonctionnait « admirablement bien ». Je me félicite donc que notre ministre fasse fonctionner admirablement bien un ministère qui fonctionne admirablement bien.

à la création d'une agence pour les TIG, les travaux d'intérêt général. Or, tout le discours que vous nous avez tenu, selon lequel les préoccupations de notre corapporteur et de la commission étaient déjà traitées par votre ministère,

l'on ne voit vraiment pas pourquoi on se poserait des questions ! Et vive les magistrats de liaison, qui réalisent, en effet, un travail très remarquable. Il n'empêche que ce que les magistrats ont dit à nos corapporteurs et aux membres de la commission des lois doit, à notre sens, être entendu.

et 200 ont obtenu une permission de sortie pour se rendre dans un bureau de vote, soit un taux d'abstention de 98 %. Pour suivre les préconisations de nos anciens collègues Jean-René Lecerf et Nicole Borvo Cohen-Seat, qui s'alarmaient de cette situation, et pour sortir de l'impasse, le présent amendement tend à mettre en oeuvre une expérimentation, afin de garantir l'effectivité du vote dans les prisons. Pour les prochaines élections européennes de mai 2019, les personnes détenues pourraient voter par correspondance, sans remettre en cause les grands principes du droit électoral- bonne information des électeurs, secret et sincérité du vote, etc. -, ni son cérémonial, avec un vote dans un isoloir prévu à cet effet. Ce dispositif serait à la fois simple, opérationnel et sécurisé, dans la mesure où les personnes détenues auraient le choix entre voter à l'urne, par procuration ou par correspondance. Le vote par correspondance existe déjà pour les Français établis hors de France ; il n'impliquerait aucune modification des listes électorales et ne concernerait que les personnes encore pourvues de leurs droits civiques ; le bon acheminement du pli serait garanti par plusieurs mécanismes de contrôle : numérotation du pli, attestation de remise, accusé de réception, etc. Le vote de cet amendement est indispensable pour organiser une telle expérimentation, le Gouvernement ne pouvant pas déroger aux dispositions législatives du code électoral. Nous mettrions ainsi en oeuvre un engagement du Président de la République, pris dans sa déclaration du 6 mars 2018 : « [ ...] On a essayé de m'expliquer pourquoi des détenus ne pouvaient pas voter, je n'ai pas compris. pas compris. Il semblerait que ce soit le seul endroit de la République où on ne sache pas organiser ni le vote par correspondance, ni l'organisation d'un bureau. La réalité, c'est que nous allons le faire et que, pour les prochaines élections européennes, je veux que tous les détenus en France puissent exercer le droit de vote ».

pour en assurer la sécurité, la faisabilité et, évidemment, la conformité juridique. Il s'agit d'instaurer une nouvelle modalité d'exercice du droit de vote pour les détenus,

force est aujourd'hui de constater que la plupart d'entre eux n'exercent pas ce droit de vote, y compris à l'occasion des grands scrutins nationaux. Le vote reste faible, voire anecdotique,

Je propose donc d'instaurer une modalité optionnelle de vote par correspondance, sous pli fermé, pour les détenus inscrits sur les listes électorales qui le souhaiteraient. Les détenus ayant choisi de voter par correspondance ne pourront dès lors plus voter à l'urne ou par procuration, mais, en cas de libération, ils pourront exercer une voie de recours devant le tribunal d'instance pour être autorisés à voter à l'urne. Une commission électorale unique, qui sera installée auprès de la Chancellerie, aura pour rôle d'établir la liste des détenus qui seront admis à voter par correspondance,

il ne sera pas possible de connaître le sens de son vote personnel. La liste des électeurs admis à voter par correspondance ne sera pas communicable, ce qui évitera toute stigmatisation des détenus. Un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application de l'article soumis à l'examen du Parlement. Il précisera, en particulier, les conditions qui permettront de garantir le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin, la composition de la commission électorale. Tel est le mécanisme que nous vous proposons,

en soit, peu importe le dispositif, il faut qu'il y en ait un ! Les chiffres avancés sont effectivement éloquents. Trop peu de détenus exercent le droit de vote, ce droit qui les relie à la cité et dont ils sont privés pour des

trouvons donc un point d'accord pour que ce droit existe et prenne corps. explication de vote. Le droit fondamental de l'exercice du vote, garanti par la Constitution, est totalement occulté en milieu carcéral, alors que les personnes sous écrou jouissent de droits civiques. Les démarches administratives sont bien trop complexes pour que les prisonniers entreprennent une procédure. Les seules solutions de rechange possibles sont le vote par procuration et les permissions de sortie, qui ne sont quasiment jamais accordées pour ce motif, et, de ce fait, pour les quelques-uns qui formulent une demande, les contraintes matérielles d'organisation entraînent des refus. Le contexte de l'incarcération représente bien un frein à l'exercice du droit de vote de la population carcérale. Comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans ses observations de 2017, seuls 2 % des personnes détenues ont pu voter aux dernières élections. Pourtant, permettre de voter au sein des prisons, c'est introduire davantage de République dans l'univers carcéral et ouvrir la voie à la réinsertion. La Pologne et le Danemark ont su implanter des bureaux de vote dans leurs prisons, sans la moindre difficulté. Ainsi souhaitons-nous saluer l'initiative présentée par le Gouvernement, même si le vote par correspondance ne permettra nullement de satisfaire la promesse formulée par Emmanuel Macron, qui s'était récemment engagé à ce que les détenus en France puissent exercer le droit de vote. Il convient donc de faire appliquer de manière effective le droit électoral des détenus, en leur offrant la possibilité de se rendre dans un bureau de vote organisé à cet effet au sein des établissements pénitentiaires. Parce qu'un vote par correspondance ne remplacera jamais l'acte consistant à mettre un bulletin dans l'urne, nous nous abstiendrons sur cet amendement.

Mme la garde des sceaux. Cet amendement vise à faire évoluer un certain nombre de dispositions législatives, pour permettre l'affectation de prévenus ayant des profils d'une sensibilité particulière et d'une réelle dangerosité dans des établissements pour peine. En l'état actuel, l'affectation de prévenus en établissements pour peine,

compte tenu de leur dangerosité. Ces dispositions ouvrent également la voie à la possibilité d'affecter des prévenus et des condamnés, indépendamment du niveau de leur peine, au sein de quartiers spécifiques spécifiques en maison d'arrêt ou en établissements pour peine. Il s'agit d'appliquer à ces prévenus ou à ces condamnés des évaluations fines et des réponses adaptées à la gestion de leur détention. Il me semble que, encadrée et circonscrite à des circonstances exceptionnelles, cette possibilité est conforme aux dispositions

publique, la loi Sauvadet, et des négociations menées avec l'État, ces cinq surveillants sont amenés à intégrer le personnel de l'administration pénitentiaire. Pouvez-vous s'il vous plaît, madame la garde des sceaux, me confirmer le calendrier prévu pour leur intégration ? Deuxièmement, la maison d'arrêt est est actuellement située dans l'enceinte de la brigade de gendarmerie, donc administrée par la garde territoriale, sous la responsabilité des gendarmes. Cette situation, qui ne devait être que provisoire, perdure depuis plus de cinquante ans. Elle ne répond pas aux standards de détention actuels, puisqu'elle ne permet ni la séparation des femmes et des mineurs, ni celle des prévenus et des condamnés. Un projet de construction d'un nouvel établissement avait été annoncé dans le courant de l'année 2016 par la Chancellerie. À ce jour, le dossier semble bloqué par vos services. Or, madame la garde des sceaux, ce dossier revêt une importance particulière, d'autant que, pour les peines d'emprisonnement supérieures à deux ans, les condamnés sont transférés à la maison d'arrêt du Camp-Est en Nouvelle-Calédonie, à plus de 2 000 kilomètres, excluant ainsi toute possibilité de visite des familles. Je ne reviens pas non plus sur la situation calédonienne, que chacun connaît, avec toutes les interrogations que cela suscite. Pouvez-vous donc, madame la garde des sceaux, me dire ce qu'il en est du projet de construction du nouvel établissement pénitentiaire à Wallis-et-Futuna ? La parole

dans sa version initiale, avant le passage en commission, prévoyait diverses mesures extrêmement dérogatoires pour accélérer les opérations d'extension et de construction des établissements pénitentiaires expropriation d'extrême urgence, enquête publique dématérialisée, etc. Madame la garde des sceaux, vous justifiez ces mesures par la nécessité de construire 7 000 places d'ici à 2022, mais, en novembre 2016, l'ancien garde des sceaux, M. Jean-Jacques Urvoas, avait déjà identifié des terrains et élaboré un plan de 15 000 places, principalement concentré sur les maisons d'arrêt et les quartiers de préparation à la sortie. Je souhaiterais savoir ce qui a été réellement prévu pour la construction de ces 15 000 places. Pourquoi la liste des implantations retenues dans le cadre de ce plan n'a-t-elle toujours pas été communiquée aux parlementaires ? Beaucoup de temps a été perdu, qui ne peut être aujourd'hui compensé par des mesures extrêmement dérogatoires et préjudiciables pour les riverains de ces établissements. Vous avez besoin de ces mesures pour accélérer les opérations de rénovation et d'extension des établissements pénitentiaires existants ... Pourquoi ne pas avoir commencé par Fresnes ? En juillet 2018, le tribunal administratif de Melun a ordonné des travaux pour l'établissement de Fresnes. de Fresnes. Il a notamment exigé un système d'évacuation d'eau et la dératisation des lieux pour cet établissement vétuste, qui se trouve dans un état épouvantable. Quelle suite a été donnée par votre ministère à cette injonction ? Peut-être, avant de promettre des places de prison, dont la programmation est aléatoire, faut-il commencer par appliquer les décisions de justice et rénover les établissements qui l'exigent De plus, comme vous le savez très bien, les dotations accordées chaque année en loi de finances pour la maintenance des établissements pénitentiaires sont insuffisantes. Les crédits dédiés à la maintenance des établissements sont régulièrement annulés en exécution.

Mais il y a des conséquences ! Le sous-investissement massif et durable dans l'entretien du parc immobilier de l'administration pénitentiaire entraîne une dégradation précoce des établissements existants et augmente les coûts de rénovation futurs. En 2017, quelque 35,7 % des cellules du parc immobilier carcéral sont considérées

Un arrêté du 8 octobre dernier a autorisé l'ouverture d'un examen professionnalisé pour ce recrutement. La date limite du retrait des dossiers de candidature est fixée au 8 novembre prochain. L'épreuve orale d'admission débutera le 15 janvier prochain. Pour ce concours,

Deux emplacements ont été identifiés : l'un sur le site de Vailepo et l'autre sur le mont Lulu. Lors d'une mission ayant eu lieu sur place, le préfet de Wallis-et-Futuna et le roi de Wallis ont fait part de leur accord sur la construction d'un

le courant du mois de septembre dernier, l'accord des autorités coutumières pour mettre le terrain à notre disposition. Il est prévu de construire un établissement de plain-pied de dix places, qui comprendra une cellule pour femme, une cellule pour mineur et huit cellules pour homme. Une dotation légèrement supérieure à 6 millions d'euros est inscrite dans le budget quinquennal à ce titre et la direction de l'aviation civile de Nouvelle-Calédonie a accepté d'assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération,

Nous avons des crédits, mais nos établissements pénitentiaires sont, pour un grand nombre d'entre eux, très anciens : il faut évidemment beaucoup d'argent pour rénover ces établissements pénitentiaires. Or, au moment où je suis arrivée 80 millions d'euros par an étaient consacrés à la rénovation des établissements pénitentiaires. Le budget pour 2019 prévoit 100 millions d'euros, et, à la fin du quinquennat, 110 millions d'euros par an seront consacrés à ces rénovations. C'est donc un engagement très fort fort que je prends, lequel suppose une programmation dans la rénovation des établissements pénitentiaires. En résumé, nous sommes bien engagés sur un programme immobilier qui comprend des constructions nouvelles, des rénovations et de la mise en sécurité sur tous les établissements.

Des promesses ont effectivement été faites, j'en ai bien conscience, et j'estime comme vous que la parole de l'État doit avoir du prix. je vous ferai observer que mon anté-prédécesseur, M. Jean-Jacques Urvoas, n'avait pas souhaité donner suite à la construction de cet établissement qui avait été envisagé sur votre territoire. J'ai moi-même pris la décision difficile de renoncer à la construction d'un établissement pénitentiaire sur votre site. Pour quelle raison ? Si j'ai pris cette décision, c'est parce que- nous venons d'en discuter -nous avons mis en place une nouvelle politique des peines qui, nous le savons, aura

ce seront 8 000 détentions en moins par an. Lorsque nous établissons les projections de population pénale,

où la projection de la population pénale ne laisse pas apparaître un besoin d'établissements pénitentiaires. Il est très difficile pour moi

? Je ne dis pas que le Président de la République n'a pas le droit de changer d'avis, et je sais que les programmes électoraux ont quelque chose de relatif. J'ai vu par le passé d'autres présidents, confrontés à la réalité des difficultés du pays, devoir renoncer à certaines de leurs propositions. Ah bon ? Ce qui me déplaît, c'est le fait de ne pas assumer un changement aussi important pour la politique pénitentiaire de notre pays. La discussion aurait pu être abordée plus facilement si cet engagement n'avait pas été pris, mais il l'a été, chacun peut le constater. Le deuxième élément pourrait venir en contrepoint de ce que je viens d'énoncer : comme je le disais tout à l'heure, le nombre de places ne peut pas à lui seul résumer une politique pénitentiaire, j'en conviens volontiers. Madame la garde des à ce qui est au coeur de votre politique, à savoir la diversification des peines. Celle-ci est nécessaire, car la sécurité de nos concitoyens ne repose pas uniquement sur l'enfermement des délinquants et des criminels pendant la durée la plus longue possible. Quand on est dans cette disposition d'esprit, on méconnaît une autre réalité : les détenus finissent toujours par sortir de prison. la politique pénitentiaire ne les prépare pas à leur sortie de prison, si elle ne comporte pas, dans le déroulement de l'exécution de la peine, une diversification des modes d'exécution de celle-ci, alors nous ne remplissons pas nos devoirs à l'égard de nos concitoyens. En effet, nous libérons une partie d'anciens détenus qui se sont endurcis et qui retombent immédiatement dans la délinquance à leur libération. D'ailleurs, l'une des grandes faiblesses du système pénitentiaire dont vous avez hérité, vous êtes là seulement depuis un an -, c'est de reposer strictement sur l'enfermement, sans que l'on ait su développer au fil des décennies à la fois le travail en prison et la diversification des modes d'exécution de la peine. Je veux bien admettre que, sur un programme de 15 000 places de prison, c'est-à-dire celui sur lequel le candidat Emmanuel Macron s'était engagé, un certain nombre de places ne correspondent pas à la vision traditionnelle que chacun se forge de la prison.

Nous aurions pu ouvrir un champ de discussion là-dessus. Et quand vous nous parlez des 7 000 places de prison au lieu des 15 000 que vous vous proposez d'achever pour 2022, madame la garde des sceaux, vous ne nous dites pas quelle est la nature de ces places ni leur ventilation entre les catégories d'établissements. J'attends avec impatience vos annonces sur tout cela.

; je ne voudrais pas que, après avoir renoncé aux 15 000 places, on en vienne en 2022 à constater que seules 3 000 places auront été ouvertes. Je rappelle que nos prisons sont actuellement occupées par près de 70 000 détenus pour un peu moins de 60 000 places disponibles, ce qui entraîne des conditions de détention parfois parfois extrêmement tendues et explique le mouvement social des surveillants de prison en ce début d'année 2018. Ce mouvement social se reproduire si des mesures ne sont pas prises, qui donnent espoir à tous nos personnels dévoués pour prendre en charge les détenus des prisons françaises.

sur le fond. Je vais effectivement présenter la carte des implantations pénitentiaires dans quarante-huit heures, à l'occasion de l'inauguration de deux établissements pénitentiaires dans le sud-est de la France. Cette carte, j'ai eu la courtoisie d'en informer l'ensemble des élus concernés, là où je projetais de construire des établissements, mais aussi là où j'avais renoncé à implanter des établissements qui avaient été précédemment annoncés : soit j'ai eu personnellement au téléphone les élus concernés, soit

Je ne ferai pas l'exégèse des textes- je m'en voudrais de m'abaisser à cela -, mais si je lis expressément le programme du président Macron, il est écrit : « Nous construirons 15 000 places de prison ».

Monsieur le président Bas, vous m'interrogez ensuite sur ce qui me semble être une question essentielle : la nature des places qui seront construites. Sur les 7 000 places de prison que nous allons livrer d'ici à 2022, nous allons en construire environ 2 000 dans des

qui permettront d'accueillir des détenus soit en fin de peine, soit en courte peine et pour lesquels il faut activement

nous devons fournir un effort extrêmement important, là encore d'ici à 2022. Par conséquent, cette diversification des établissements entre maisons d'arrêt, centres pénitentiaires à régimes diversifiés, structures d'accompagnement vers la sortie nous permet d'accueillir les détenus selon

en faveur de l'activité des détenus en termes de formation, mais également de travail. J'ai commencé à nouer un dialogue avec ma collègue Muriel Pénicaud

différenciées, que cette gamme d'établissements pénitentiaires nous permettra d'accueillir les personnes condamnées en fonction de la nature de leur peine, de leur dangerosité, de leur parcours

Je souhaite que la diminution de la population carcérale résulte de la politique des peines que nous avons construite et que j'aurais aimé vous voir voter. C'est bien parce que la politique des peines que je propose

dans les meilleures conditions. C'est aussi la raison pour laquelle je propose, outre des peines alternatives à la prison, des peines autonomes, qui seront sans lien avec la prison.

est largement avancée et qu'apparaissent des difficultés tout à fait localisées susceptibles de retarder l'exécution. Les mesures contenues dans l'article 51, dont celle-ci, sont à mes yeux indispensables pour que nous puissions disposer, dans les délais que nous nous sommes fixés, des établissements pénitentiaires dont nous avons besoin. monsieur le rapporteur,